Or, avec une inflation excessivement faible, il n'y aura pas de soutien au pouvoir d'achat des Français, qui réclament aujourd'hui davantage de justice sociale et fiscale, c'est-à-dire une meilleure redistribution des richesses. L'article 2, tel qu'il est rédigé, n'est pas à la hauteur de la question sociale. monsieur le ministre : la pauvreté augmente dans notre pays. Lisez par exemple le rapport de France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon, qui a repris avec près d'un an de retard les conclusions d'un rapport que j'avais commis avec l'ancien rapporteur général de

Depuis le début du quinquennat, les élus de gauche vous alertent sur les conséquences socio-économiques de votre politique fiscale. Vous avez ignoré à maintes reprises ces mises en garde. Les élus socialistes de cette chambre vont donc proposer par voie d'amendement des mesures fiscales ambitieuses pour contribuer à une meilleure redistribution des richesses dans notre pays. En effet, avec le simulateur LexImpact, mis à notre disposition, nous avons réussi à mieux répartir l'impôt sur le revenu sans porter atteinte aux recettes de l'État, afin de renforcer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. À l'heure actuelle, la situation économique du pays est préoccupante. On compte 800 000 emplois supprimés en 2020, un million d'individus tombés dans la pauvreté et une multiplication de plans sociaux- Nokia, Sodexo, Airbus, etc. -, le tout en l'espace de quelques mois. Et le confinement deuxième du nom ne sera pas sans conséquence. Pendant que le pays s'effondre, vous continuez à défendre avec vigueur les intérêts d'une classe, celle des très très très riches. La situation impose que les très hauts revenus soient mis à contribution pour participer à l'effort de guerre.

! Après un grignotage de 5 milliards d'euros- ce n'est tout de même pas une petite affaire -, vous retranchez de nouveau le produit de cet impôt essentiel. Nous vous proposons, en passant à onze tranches, une mesure de justice fiscale, afin que chacun paye un impôt au plus près de ses revenus ses revenus et de ses ressources. Vous nous direz peut-être, comme nous l'avons entendu ces dernières années, que cette proposition est « confiscatoire ». Aujourd'hui, 45 % sont prélevés pour la fraction des revenus supérieurs à 158 122 euros. Nous souhaitons une augmentation de dix points.

est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Yves Leconte. L'alinéa 15 de l'article 2 du présent PLF pour 2021 ajuste en fonction des 0,2 % d'inflation les montants retenus pour la réforme de la décote devant entrer en vigueur le 1 janvier 2021 et applicable aux revenus perçus en 2020. Cette réforme était issue de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Elle a donc été adoptée avant la pandémie et la crise sanitaire liée au covid-19, que toutes et tous ont eu à subir au cours de cette année,

que le Gouvernement avait proposée au début de l'année 2020. Cette baisse, de 5 milliards d'euros au total, portait principalement sur les deux premières tranches. Ce sont ainsi 17,5 millions

« La crise a exacerbé les inégalités de revenus ». La situation ne fait qu'empirer, d'où l'urgence impérative d'une meilleure progressivité de l'impôt.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

sur le texte qui avait été voté en 2019, sans concertation aucune, pour abaisser le plafond d'abattement sur l'impôt sur le revenu.

soit une donnée réelle dans notre République, et non pas un espoir pour tant de gens qui ne se sentent pas respectés en tant que citoyens. Effectivement, nombreux sont ceux et celles qui ne payent pas l'impôt sur le revenu,

Cet amendement vise à soustraire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants. Aujourd'hui, le mal-logement concerne en France 3,8 millions de personnes. En parallèle, 12 millions de personnes sont fragilisées s'agissant du logement et se retrouvent proches d'une situation de mal-logement impayé de loyer, effort financier excessif, copropriété en difficulté, précarité énergétique, surpeuplement modéré ... Parmi ces personnes, 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12 % par rapport à 2015.

De plus, malgré les efforts mobilisés par plusieurs gouvernements pour la construction de nouveaux logements sociaux, le temps moyen pour obtenir un logement n'a cessé d'augmenter, notamment en raison de la réticence de certains maires qui refusent de construire. Pour les baux signés en 2019, la durée moyenne entre la demande de logement social et la signature du bail s'établit en moyenne à trente-trois mois en Île-de-France, contre trente et un en 2018. Pour lutter efficacement contre la crise du logement tout en continuant les programmes engagés, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires privés de biens immobiliers. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Je ne suis

Aujourd'hui, il existe un conflit entre la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'État. La doctrine administrative considère que la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires

en proposant que les rémunérations des fonctions techniques des associés des sociétés d'exercice libéral soient traitées fiscalement comme des traitements et salaires.

Sous la mandature précédente, l'exonération d'impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour enfant élevé ou à charge a été supprimée à compter de l'imposition des revenus de 2013 alors qu'elle existait depuis 1941. Le Gouvernement motivait cette décision par le fait que c'était essentiellement les pensions les plus élevées qui bénéficiaient de cet avantage fiscal. L'intégration de la majoration de pension dans le calcul de l'impôt sur le revenu a rendu en réalité de nombreux retraités modestes imposables. Le présent amendement a pour objet de rétablir l'exonération. En effet, sa suppression a conduit à une augmentation de l'impôt sur le revenu pour un grand nombre de foyers fiscaux et à en faire entrer certains dans l'impôt sur le revenu alors qu'ils n'étaient pas imposables. Il est donc proposé de rétablir l'exonération d'impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour enfant élevé ou à charge.

est à Mme Laure Darcos. Le 9 juillet 2018, à l'occasion de son discours devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République avait annoncé l'inscription d'une réforme du grand âge et de l'autonomie au programme de travail du Gouvernement pour 2019. En 2050, la France comptera près de 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui ne pourront plus se lever ou faire leur toilette seules, préparer ou prendre un repas sans dépendre d'autrui. Nombre de personnes âgées seront aussi sujettes à des altérations de la mémoire.

parce qu'elle est deux fois plus élevée que la statistique qui fait foi dans les rapports officiels et qui figure dans les documents du ministère de la santé et des solidarités. Dans ce contexte, nous devons penser aux aidants. En France, entre 8 millions et 11 millions d'aidants soutiennent un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Ce dévouement solidaire se fait parfois au détriment de la vie personnelle, sociale et professionnelle du proche aidant. C'est pourquoi, au surplus d'autres mesures qui ont été ou devront être mises en place pour affronter ce défi, il est ici proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu les ressources de l'allocation personnalisée d'autonomie employées pour rémunérer un proche aidant. Il s'agit d'une mesure en faveur de la solidarité intergénérationnelle, solidarité d'autant plus nécessaire en période de crise. Tel est le sens de cet amendement, auquel j'associe particulièrement notre collègue Jocelyne Guidez, qui est très active sur ces questions. Quel est l'avis de la commission

Ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu depuis la loi de financement sur la sécurité sociale pour 2020. En fait, le dispositif proposé prévoit de cumuler deux dispositifs d'aide pour que le salaire perçu par le proche aidant et financé par le biais de l'APA

Depuis le début du premier confinement, nos concitoyens sont confrontés à une très forte augmentation du coût de la vie- mise en place du télétravail, coût des masques et des mesures barrières dans les trajets domicile-travail -, qui demeure pour partie à leur charge, malgré les dispositifs existants. Bien que les contribuables soient autorisés à déduire de leurs revenus les frais professionnels supplémentaires dans le cadre d'une option pour les frais réels, option admise sur l'initiative du contribuable, le contexte très particulier de cette année va exclure du dispositif de nombreux Français, car la priorité est d'abord sanitaire avant d'être comptable. Le présent amendement vise à assurer une forme de justice sociale et d'équité fiscale, en augmentant temporairement le taux forfaitaire d'abattement pour frais professionnels, qui est légalement fixé à 10 % des revenus, à 25 %, afin de prendre en compte les nombreux frais induits, qui sont nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle dans cette période particulière. L'option pour les frais réels demeurerait possible pour les contribuables qui le souhaiteraient.

Certaines catégories de contribuables sont plus fragiles que d'autres et doivent donc faire l'objet d'une protection particulière. C'est le cas des personnes âgées de plus de 65 ans et de celles qui sont frappées d'invalidité. Ne pouvant plus bénéficier de revenus du travail et étant placées dans une situation de dépendance au regard de la politique de revalorisation des pensions et des allocations, une protection fiscale particulière doit leur être accordée. Un abattement spécifique existe déjà, mais il est considéré comme trop faible, compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat des retraités depuis le début du quinquennat. Ainsi, la dernière étude de l'Insee disponible sur ce sujet, qui date de mars 2019, estime que, alors qu'entre janvier et octobre 2018 le niveau de vie de l'ensemble des Français a baissé de 0,4 % en moyenne, celui des retraités a baissé, lui, de 2 %, soit un écart de 1,6 point. Il est donc proposé de doubler le plafond des abattements spécifiques prévus pour ces contribuables. la sénatrice, vous évoquez la chute du pouvoir d'achat des retraités depuis le début du quinquennat. Je ne suis pas sûr néanmoins qu'elle doive entraîner un doublement de l'abattement spécifique qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans.

présenter l'amendement déposé par Mme Boyer, j'ai reconnu l'exposé des motifs. L'affirmation sur l'évolution du pouvoir d'achat des retraités à l'échelle du quinquennat

s'il était voté, d'assurer une période de transition, durant laquelle le foyer fiscal qui disposait d'au minimum deux parts bénéficierait temporairement d'un minimum d'une part et demie, avant de revenir à un régime d'une part. part. Les ménages les plus modestes se trouvent doublement touchés par ce drame familial : ils se voient immédiatement affectés par la perte d'un avantage fiscal acquis lors de l'union civile contractée

La réintroduction de la demi-part sans distinction, entreprise par l'ancienne majorité parlementaire en 2014, n'est pas souhaitable. Il s'agit en effet d'un dispositif trop coûteux et qui ne cible pas les ménages qui en ont réellement besoin, en raison de la précarité de leur situation. L'objet de cet amendement est donc la mise en place d'un dispositif d'aide aux ménages ayant connu la perte d'un conjoint ou d'une conjointe. Cette mesure ne saurait être généralisée : son objectif est de sécuriser les ménages les plus modestes.

soumis à l'impôt séparément de leur père ou de leur mère. Ce dispositif bénéficiait également aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés. Désormais, seuls les parents isolés ayant eu effectivement un ou plusieurs enfants à charge peuvent prétendre à la demi-part supplémentaire sous conditions. Je vous rappelle néanmoins que des mesures ont été prises pour compenser les hausses d'impôts subies par les personnes veuves. Ainsi, depuis 2018, l'éligibilité à l'impôt de veufs ou de veuves ne bénéficiant pas, dans le nouveau système, de la demi-part dont ils bénéficiaient auparavant ne les conduit plus à être assujettis à certains impôts locaux, comme la taxe d'habitation.

un ascendant en perte d'autonomie. Il s'agit d'une mesure en faveur de la solidarité intergénérationnelle, solidarité d'autant plus nécessaire en période de crise.

à porter à 1 000 euros la réduction d'impôt sur le revenu au titre des revenus 2020 pour les dons faits aux associations d'aide aux personnes en difficulté. Dans la période actuelle de crise sanitaire, bon nombre de nos concitoyens

mais cette mesure ne concerne pas les donateurs non imposables, dont le nombre était pourtant estimé à 21,4 millions en 2017.

pas déjà, je précise qu'il s'agit de mettre en cohérence ce projet de loi de finances avec l'article 4 de la loi de finances rectificative, qui a relevé le plafond de non-imposition à 7 500 euros pour les heures supplémentaires réalisées pendant l'état d'urgence par les personnels médicaux. Il s'agit d'étendre ce dispositif au temps de travail additionnel. Quel

l'avis du Gouvernement ? Le coût serait important, mais je ne peux le chiffrer au moment où je m'exprime. L'avis est défavorable, en cohérence avec les positions exprimées lors des débats sur le PLFR 2 et le PLFR 3, alors que le président Karoutchi avait déjà déposé des amendements analogues. Nous considérons que, avec l'exonération plafonnée à hauteur de 5 000 euros, 94 % des salariés qui réalisent des heures supplémentaires sont couverts. En portant ce plafond à 7 500 euros

tenir compte de la politique de la France en faveur de la transition énergétique, il paraît opportun de pouvoir adjoindre les travaux dits de rénovation énergétique à ce dispositif

types d'avantages sur les mêmes dépenses. Par ailleurs, il y a une position constante qui consiste à considérer que les travaux d'amélioration énergétique, et donc de rénovation, des locaux à usage professionnel sont aussi des facteurs d'augmentation de la valeur du bien. Ils n'ont pas la même finalité ni la même

des articles non rattachés, vous trouverez une disposition adoptée à l'Assemblée nationale, à la suite d'un amendement proposé par le Gouvernement, qui crée, à titre temporaire, un crédit d'impôt au bénéfice des PME dans le cas de la rénovation énergétique des bâtiments

de particuliers propriétaires de locaux commerciaux et professionnels, donc ils ne seront pas non plus concernés, alors même que l'objectif de l'avantage fiscal institué par le Gouvernement en seconde partie rejoint exactement la préoccupation que je suis en train d'exprimer ici pour les particuliers propriétaires de locaux. Soit la rénovation énergétique est une politique prioritaire de notre pays tendant à réduire la consommation d'énergie et à stimuler l'économie, soit on empile des dispositifs qui ne sont pas cohérents. Moi, j'essaie d'être cohérent

M. Didier Marie. À l'heure où le Gouvernement prône un virage écologique, cet amendement vise à promouvoir l'économie circulaire dans les achats quotidiens des Français, en proposant la création d'un crédit d'impôt de 50 % pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques, informatiques, ainsi que sur les bicyclettes, les chaussures et produits en cuir, l'ameublement, les vêtements et le linge de maison, et ce dans la limite de 2 500 euros par foyer fiscal.

l'économie circulaire, à laquelle nous aspirons tous.

Au risque de la contradiction avec ce que je viens de dire sur le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des PME, le Gouvernement est généralement assez peu favorable, c'est un euphémisme, à la création de dépenses fiscales et de crédits d'impôt. C'est donc un avis défavorable sur les deux amendements.

Cette disposition répond à deux nécessités : d'une part, conforter les fonds propres des coopératives en rendant plus attractive la souscription de capital social ; d'autre

Cependant, exonérer d'impôt les produits de cession et les intérêts qui rémunèrent des parts sociales me semble aller trop loin au regard du principe d'égalité devant l'impôt. Il convient en effet de rappeler que les acquisitions de parts sociales

M. Vincent Segouin. Les intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes ont conduit à la constatation de l'état de catastrophe naturelle pour cinquante-cinq communes. Les dégâts matériels sont immenses.

par des organismes volontaires qui sont aujourd'hui exclus du dispositif. Je rappelle que la commission des finances avait émis l'an passé un avis favorable à une telle ouverture, lors de l'examen du projet de loi de finances pour

M. Emmanuel Capus. Comme vous le savez, le secteur du sport professionnel se trouve actuellement dans une situation dramatique, du fait de la crise sanitaire, parce que les recettes des clubs ont énormément baissé faute de billetterie. Dans ce contexte, nous devons renforcer l'attractivité de la France comme terre de champions, notamment dans la perspective des jeux Olympiques de 2024. C'est pourquoi je défends cet amendement, déposé par notre collègue Joël Guerriau, vise à renforcer la France comme terre d'attractivité pour les talents sportifs. Concrètement, cet amendement tend à maintenir le régime de l'impatriation lorsqu'un sportif professionnel change de club au sein d'un même championnat sportif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui : dès qu'il change de club, il perd son régime. Il s'agit d'utiliser le même régime fiscal que celui des cadres étrangers rejoignant des entreprises françaises.

est l'avis du Gouvernement ? Le maintien du régime des impatriés en cas de changement de club favoriserait la mobilité des seuls sportifs professionnels recrutés à l'étranger, ainsi que la mobilité des sportifs professionnels en dehors de leur club d'origine, ce qui nuirait aux clubs qui ont pris le risque de les faire venir en France. Par ailleurs, il ne nous paraît pas qu'un motif d'intérêt général puisse justifier que des sportifs professionnels recrutés en France dans des conditions de droit commun conservent le bénéfice d'un régime fiscal de faveur dont le seul objectif est de favoriser le recrutement à l'étranger des talents nécessaires à la vie de la Nation. Pour ces raisons, l'avis du Gouvernement

ce sans risquer de redressement fiscal. Certaines exploitations agricoles ont été sévèrement impactées par la crise sanitaire, qui a entraîné une diminution des ventes, laquelle se répercute sur la récolte de l'année 2020. Dans ces conditions, certains loyers fixés avant la crise apparaissent désormais difficilement supportables. Il ne s'agit pas d'obliger les bailleurs à réduire leurs loyers, mais de permettre à ceux qui en ont les moyens d'accepter une diminution de loyer, temporaire ou plus durable, par avenant au bail initial, sans risque de redressement fiscal. Ce dispositif serait néanmoins encadré, le nouveau fermage devant s'inscrire dans le cadre des fourchettes fixées par arrêté préfectoral, conformément au code rural. Le coût budgétaire d'une telle mesure serait limité, dès lors que la diminution des revenus des bailleurs sera compensée par une amélioration des résultats imposables des entreprises.

comme un outil pédagogique pour apprendre aux gens à boursicoter, ce qui est une excellente idée ... À voir ... rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, avait défini ce système comme un « trou noir fiscal » dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2020. Cette dépense fiscale n'a pas pour fondement un dispositif législatif, mais une simple instruction,

l'imposition, nulle exonération d'imposition ne s'applique, dès lors que ces gains sont imposés au niveau des adhérents à l'occasion de leur retrait ou de la dissolution du club d'investissement. Le seul avantage réside dans le différé d'imposition, qui tient au réinvestissement immédiat par le club

concurrence des marchés étrangers, très fortement concurrentiels en raison de la réforme des fiscalités. La conséquence en est directe : bon nombre des livres imprimés en langue française et vendus en France sont désormais imprimés à l'étranger. Aussi, afin de permettre aux imprimeries implantées en France de conserver leur rôle historique d'impression, mais également les emplois qu'ils créent dans les territoires, il convient de leur octroyer

imprimeurs implantés en France et respectant un nouveau label intitulé « Imprimerie éco.citoyenne », mis en place par l'autorité administrative, qui porterait sur trois points : le respect de l'environnement, les efforts pour la maîtrise des consommations d'énergie et la protection de la filière bois.

Cet amendement concerne les non-résidents dits « Schumacker », établis dans les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Ces contribuables tirent de la France l'essentiel de leurs revenus imposables. Le régime fiscal qui leur est applicable découle d'un arrêt du 14 février 1995 par lequel la CJUE CJUE a jugé qu'un État membre a l'obligation de traiter à l'identique les non-résidents et les résidents, lorsque les premiers se trouvent dans une situation comparable à celle des seconds du fait qu'ils tirent de l'État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Le régime Schumacker s'applique également aux personnes fiscalement domiciliées en Suisse qui tirent d'un État membre l'essentiel de leurs revenus, et ce en vertu de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes. La jurisprudence Schumacker a été reprise par la doctrine administrative fiscale. Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, je vous propose de la faire figurer dans le code général des impôts. Je vous propose également de faciliter le recours au régime Schumacker, en permettant aux contribuables concernés d'en solliciter l'application en annexant à leur déclaration de revenus une déclaration sur l'honneur. Cette proposition s'inspire directement d'un rapport que le Gouvernement a récemment remis au Parlement.

dont la quasi-totalité des revenus sont de source française et qui ne bénéficient pas de mécanismes de nature à réduire leurs impôts dans leur pays de résidence, d'être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France. Ils peuvent ainsi bénéficier de réductions d'impôt ou de crédits d'impôt, contrairement au reste des non-résidents fiscaux. Le critère de domiciliation crée forcément des inégalités fiscales entre les différentes catégories de non-résidents. catégories de non-résidents. Cet amendement vise à permettre aux personnes résidant dans un État tiers qui a conclu une convention bilatérale avec la France comportant un échange d'informations fiscales,

Cet amendement a pour objet de permettre la déductibilité des charges supportées par tous les non-résidents, y compris ceux qui sont établis dans les États tiers à l'Union européenne autres que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, qui, d'une part, tirent l'essentiel de leurs revenus de la France et, d'autre part, ne bénéficient dans leur État de résidence d'aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale. Actuellement, seuls les non-résidents Schumacker peuvent de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.

je veux préciser que cette jurisprudence Schumacker s'impose à tous les États membres, mais que cette réciprocité n'est pas possible entre la France et un pays tiers. En clair, un Français non résident dans un autre État ne bénéficie pas des mêmes avantages.

qui vivent dans des zones particulièrement dangereuses et qui ont besoin de conserver une habitation en France. est défavorable à cet amendement, qui vise à assimiler la résidence détenue en France par un contribuable non résident à sa résidence principale, lorsqu'il réside dans une zone déconseillée aux voyageurs.

D'autre part, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts, la résidence principale entraîne la domiciliation fiscale en France,

plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des non-résidents fiscaux, ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas lorsque le cédant est une personne morale comme une SCI, alors même que, pour les résidents, l'exonération est possible lorsque la SCI a été mise à la disposition gratuite de l'un des associés à titre de résidence principale. Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux associés non-résidents d'une SCI. Je sollicite l'avis du Gouvernement sur cet amendement, qui vise à exonérer les plus-values de cession pour les biens cédés par un associé non résident d'une SCI. SCI. Je suis plutôt réticent à un nouvel élargissement du dispositif pour y inclure les associés non-résidents d'une SCI, car vous créez ainsi une inégalité de traitement qui ne paraît pas justifiée.

est une disposition propre aux non-résidents, mise en oeuvre par la loi de finances pour 2014. Elle leur permet de céder de manière particulièrement dérogatoire un logement libre d'imposition sur les plus-values, alors même qu'il ne constituait pas leur résidence principale en France. Par conséquent, votre proposition reviendrait à avantager encore un peu plus ces derniers par rapport aux contribuables résidents, ce qui est discutable au regard du principe d'égalité devant l'impôt. Je tiens aussi à souligner que, s'agissant de la cession de leur ancienne résidence principale en France, les non-résidents ont déjà été mis sur un pied d'égalité avec les résidents par la création de dispositions spécifiques à l'article 244 A du code général des impôts, qui n'impose d'ailleurs pas comme condition

a été votée dans la loi de finances pour 2019. Cette réforme n'avait fait l'objet d'aucune concertation avec l'ensemble des élus des Français de l'étranger ni d'une étude d'impact exhaustive, dont le Parlement aurait pu disposer pour éclairer ses votes. Très vite, nos compatriotes, les sénateurs, les conseillers consulaires et les associations des Français de l'étranger ont dénoncé des effets de bord, voire des effets confiscatoires, des augmentations d'impôt de 20 % à 400 %. Un moratoire a dû être adopté dans la loi de finances pour 2020. Un rapport du Gouvernement au Parlement a démontré le bien-fondé des protestations de nos compatriotes non-résidents. L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à abroger cette réforme pour revenir au régime antérieur. Néanmoins, un élément de la réforme fiscale de 2019 subsiste : l'augmentation du taux minimum d'imposition à 30 % pour la fraction des revenus supérieure à 27 519 euros. Nous avons déposé plusieurs amendements de suppression de ce dispositif lors de la discussion des derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat a adopté à plusieurs reprises, les 27 novembre 2018 et le 23 novembre 2019

le rapporteur et dont l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale n'est pas programmée. Nous proposons donc de faire revoter un amendement similaire à ceux qui ont été votés par le Sénat pour revenir définitivement et complètement sur la réforme fiscale des revenus de source française des non-résidents, particulièrement de nos compatriotes expatriés.

Monsieur le ministre, qui consistait à supprimer le caractère libératoire de la retenue spécifique à la source appliquée à ces revenus. D'ailleurs, il faut souligner que nous parlons non pas de contribuables non-résidents, mais bien de revenus non-résidents, puisque certains contribuables résidant en France peuvent percevoir des revenus considérés comme non-résidents, et inversement. Le Gouvernement a aussi estimé que les premières étapes de la réforme de l'imposition des revenus non-résidents étaient justes, parce qu'elles garantissent une meilleure progressivité du système d'imposition. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l'amendement présenté par Mme la sénatrice Deromedi.

de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu'elles sollicitent l'application du taux moyen d'imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu'elles n'ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence. Dans un souci de cohérence, je propose d'autoriser la déduction des prestations compensatoires qui sont imposables en France. Je rappelle qu'une disposition allant dans le même sens a récemment été adoptée par notre assemblée à l'occasion de la discussion d'une proposition de loi relative aux Français établis hors de France. L'amendement

les pensions alimentaires aux prestations compensatoires. qui visent à permettre aux non-résidents imposés au taux moyen de déduire de leur revenu imposable les prestations compensatoires consécutives à un divorce. Dans la mesure où ces prestations compensatoires sont généralement liées au versement d'une pension alimentaire et où le taux moyen prend en compte la situation familiale des non-résidents, cette demande ne me paraît pas illégitime.

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier de la décote. Contrairement aux non-résidents Schumacker, les contribuables établis dans les États tiers de l'Union européenne, autres que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la France ne peuvent pas bénéficier de la décote. Une telle différence de traitement est à mon sens contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Elle a pour effet d'exclure de la baisse de l'impôt sur le revenu des personnes qui ont aussi contribué au redressement de nos finances publiques. En droit, rien ne s'oppose à ce que tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère soient placés sur un pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter le présent amendement.

spécifique sur les revenus des non-résidents, et du fait de son caractère libératoire, l'assiette imposable des non-résidents est considérablement réduite. Il ne paraît pas justifié, dans ce contexte, de leur étendre le bénéfice du mécanisme de la décote. le bénéfice de la décote s'appliquerait, dans votre système, à l'ensemble des contribuables non-résidents déclarant des revenus de source française, quelle que soit leur nature, c'est-à-dire à ceux qui perçoivent des revenus ou des pensions, mais également à ceux auxquels on verse des revenus fonciers, par exemple. Enfin, le rapport du Gouvernement au Parlement sur la fiscalité appliquée aux revenus des non-résidents explique qu'un tel dispositif donnerait un avantage excessif aux non-résidents. Pour toutes ces raisons,

il tend à rembourser l'intégralité des frais de scolarité des enfants des non-résidents scolarisés dans un établissement français de l'étranger. Les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient certes d'une réduction d'impôt, mais celle-ci est bien moindre.

n° I-142 rectifié. Nous proposons l'extension aux non-résidents et, par conséquent, à nos compatriotes expatriés de la réduction d'impôt pour dons aux oeuvres, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. Le refus d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts est une réelle source d'incompréhension pour les Français non-résidents. Les versements au profit de ces organismes permettent à nos compatriotes de garder un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères, les initiatives associatives venant souvent pallier l'insuffisance des interventions publiques et nécessitant pour cette raison des soutiens financiers stables et récurrents. le Sénat a déjà adopté cette disposition sur l'initiative de la commission des finances dans le cadre de la proposition de loi relative aux Français de l'étranger, présentée par M. Bruno Retailleau et dont

les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas de déductions de charges et de crédits d'impôt. Ils ne peuvent donc pas défiscaliser les dons qu'ils consentent aux organismes d'intérêt général. Cet amendement vise à ouvrir cette possibilité à une catégorie particulière de dons, ceux qui sont effectués à des établissements à des établissements scolaires du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour leurs projets de développement et de rénovation. Cette disposition, par sa dimension incitative, contribuerait à atteindre l'objectif fixé à l'origine par le Président de la République, qui est le doublement du nombre des élèves dans les lycées français à l'étranger d'ici à 2025, surtout dans un contexte de fragilisation du réseau en raison de la crise.

Cette réduction d'impôt serait égale à 100 % du montant des sommes versées, soit une déductibilité totale de ces dons. Sans plafond, sans rien ? C'est une incitation forte à aider ces acteurs de la solidarité dans le contexte que nous connaissons. Ils incarnent, évidemment, le troisième pilier de la devise républicaine : la fraternité. Quel est l'avis de la commission Je demande le retrait de cet amendement, au profit de celui qui sera déposé en deuxième partie de ce texte.

Je suis profondément défavorable à l'amendement n° I-199 rectifié, dont je mesure- et il faut que vous le mesuriez aussi, monsieur Temal -qu'il pourrait avoir des conséquences assez néfastes, pour ne pas dire plus, sur le fonctionnement de la vie politique française.

Par crainte que la même chose ne se produise pour trois autres prélèvements, à savoir le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, le Gouvernement les a alors fusionnés et a introduit un nouveau prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % affecté directement au budget de l'État.

tout en continuant à faire contribuer à l'impôt l'ensemble des contribuables disposant de revenus patrimoniaux de source française. Exonérer les non-résidents créerait une différence de traitement que je considère comme injustifiée.

Il a pour objet d'exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour.

Le problème est simple. Contrairement aux ressortissants d'États tiers mariés à un citoyen non français, comme, par exemple, un Indien qui aurait épousé une Belge, les les conjoints extracommunautaires de Français doivent s'acquitter d'une taxe au moment de la délivrance ou du renouvellement de leur carte de séjour. Autrement dit, ceux qui ont épousé un Français sont pénalisés par rapport à ceux qui ont eu cette chance, en quelque sorte, de ne pas en avoir épousé un. Comme je l'ai dit, le Défenseur des droits a souligné à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une « discrimination à rebours fondée sur la nationalité mes chers collègues, à mettre fin à cette discrimination inacceptable. Je propose également de rendre gratuite la délivrance d'un duplicata pour les conjoints étrangers de Français, les conjoints étrangers de Français victimes de violences conjugales

vous le savez, mes chers collègues, des exemptions sont déjà prévues pour la primo-délivrance du titre de séjour, quand cela est justifié. Elles visent notamment les étrangers protégés et vulnérables, ceux qui relèvent d'accords internationaux, c'est-à-dire

Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas négligeable.

de la carte du combattant ou de la pension militaire d'invalidité, indépendamment de l'âge de décès de ce dernier. Sur l'initiative de nos collègues députés,

Les plans d'épargne retraite populaire ont vocation à être transférés dans des plans d'épargne retraite, selon le nouveau dispositif issu de la loi Pacte. Le présent amendement vise à assurer la neutralité fiscale des transferts d'actifs qui vont intervenir

Mme Isabelle Briquet, sur l'article. L'article 3 du présent projet de loi de finances baisse la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à hauteur de la part affectée aux régions et ajuste le le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée. Baisser les impôts de production, pourquoi pas ? Ah ? Mais cela ne peut se faire sans condition, que ce soit en termes d'emploi ou d'investissement. Le ministre de l'économie prétend avoir demandé des contreparties, mais vous semblez seulement compter sur le bon vouloir des entreprises- possible, mais très incertain. Surtout quand le Medef salue dans un communiqué, le 28 septembre dernier, les « mesures destinées à renforcer les fonds propres des entreprises Monsieur le ministre, en ces temps de crise, plutôt que de satisfaire le patronat, plutôt que de renforcer les fonds propres des entreprises, ne faudrait-il pas les obliger à investir dans la transition écologique ? Ne faudrait-il pas les obliger à investir dans l'emploi des jeunes ? Avec cet article 3, vous faites un chèque en blanc aux actionnaires du CAC 40. Bah voyons ! En effet, la CVAE, qui est notamment visée par cette baisse, concerne les seules entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 000 euros. Ainsi, cette baisse des impôts de production ne profite aucunement aux TPE et très peu aux PME. Vous privilégiez une nouvelle fois les grandes entreprises plutôt que les TPE-PME.

: le financement du contrat de présence postale. La réforme que vous engagez aura un impact direct et négatif sur le financement de la mission d'aménagement du territoire confiée au groupe La Poste. Cette mission, vous le savez, permet d'assurer un maillage territorial postal le plus dense possible sur l'ensemble du territoire. Pour assurer le financement de cette présence postale, un Fonds postal national de péréquation territoriale est alimenté par un abattement sur la taxe locale due par La Poste, touchant essentiellement la Le montant de ce fonds s'élève à 174 millions d'euros en 2020. La réforme fiscale engagée devrait entraîner une diminution substantielle du montant de ce fonds, de l'ordre de 65 millions d'euros, en 2021 et en 2022. Cette perte doit donc être compensée pour permettre la poursuite des actions menées par les 100 commissions départementales de présence postale territoriale. Ces actions en faveur des zones rurales, des zones de montagne, des quartiers de la politique de la ville et des départements ultramarins, nous les considérons comme prioritaires et totalement indispensables. Le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises a indiqué à l'Assemblée nationale, le 7 novembre dernier, que des discussions étaient en cours au ministère de l'économie et des finances pour trouver une solution permettant de maintenir le niveau actuel du fonds de péréquation postale à hauteur de 174 millions d'euros et maintenir ainsi le niveau de financement de la mission d'aménagement du territoire de La Poste à cette même hauteur.

approuvons ces mesures, car il est vraiment nécessaire, aujourd'hui, d'aider nos entreprises à être beaucoup plus compétitives et de les mettre sur un pied d'égalité avec les autres entreprises de l'Union européenne.

des analyses menées en relation avec cet article, 75 % de la baisse d'impôt que nous proposons bénéficiera aux PME et aux ETI. C'est notre volonté politique que d'accompagner plus fortement ces catégories d'entreprises, considérant qu'elles participent directement à tout ce qui relève de la relocalisation, mais aussi, pleinement, à la création d'emploi sur les territoires. C'est dans cette catégorie d'entreprises que les créations d'emplois sont les plus nombreuses. Troisièmement, je veux souligner que

15 % à la filière du transport, de l'entreposage et de la logistique, de 15 % au commerce, le reste se répartissant sur l'intégralité des filières.

la réduction de la participation des entreprises à ce qui fait le contrat social, à ce qui fait nos services publics, à ce qui fait aussi la France. Je pense que cela ne va pas dans le bon sens.

Le Gouvernement nous vend la nécessité de combler un différentiel de compétitivité, notamment par rapport à l'Allemagne, où les impôts dits « de production » seraient moins

Ce remplacement de la fiscalité locale par une dotation est une forme de tutelle, ni plus ni moins, les dotations pouvant évoluer à la baisse dans la durée. Après la suppression de la taxe professionnelle en 2010, celle de la taxe d'habitation et maintenant celle, lancée, d'une partie significative des impôts des entreprises,

Si les États ne parviennent pas à reprendre la main et à retrouver une capacité à taxer les profits des entreprises, alors le financement de notre modèle social reposera de plus en plus sur les ménages et la lutte contre les inégalités n'en sera que plus difficile.

en pleine période de covid. D'habitude, le capital coûte 200 milliards d'euros par an en France, à travers 6 000 dispositifs. Cette année-

Le scrutin est ouvert.